Monsieur le président,

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 9 février 2017 sur les contrôles et les sanctions en matière de concurrence en Polynésie française qui s'est réunie Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, c'est-à-dire sans habilitation du Parlement, de sorte qu'elle doit être expressément ratifiée dans un délai de dix-huit mois, sous peine de caducité. Ce délai expire le 10 août prochain. Cette ordonnance prévoit principalement les voies de recours contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence et les prérogatives d'enquête de cette autorité pouvant affecter les libertés publiques, en matière de pratiques anticoncurrentielles. Ces deux matières relèvent de la compétence du législateur national, qui a complété ici des dispositions déjà adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française, laquelle a décidé en 2014 de se doter d'un code de la concurrence, inspiré du livre IV du code de commerce national, et de créer une autorité polynésienne de la concurrence, sur le modèle de l'Autorité de la concurrence métropolitaine. La détermination des prérogatives et des pouvoirs d'enquête ordinaires de l'Autorité polynésienne de la concurrence relève de la compétence de l'Assemblée de la Polynésie qui a d'ailleurs adopté il y a quatre mois, le 14 mars dernier, une nouvelle loi du pays pour modifier certains aspects du code de la concurrence et des missions de l'autorité. Avec la ratification de cette ordonnance, nous venons donc conclure ce processus d'élaboration d'un droit moderne de la concurrence en Polynésie. Madame la ministre, il nous faut malheureusement constater que ce processus aura été particulièrement long écoulés depuis l'adoption de la première loi du pays en juin 2014 ! Que de temps perdu, mes chers collègues, alors que l'Autorité polynésienne de la concurrence a été officiellement installée en février 2016 En novembre 2014, l'Assemblée de la Polynésie française a demandé à l'État de prendre les dispositions complémentaires relevant de sa compétence. Le projet d'ordonnance n'a été transmis à l'Assemblée de la Polynésie française qu'à la fin de l'année 2016, soit deux ans plus tard. L'ordonnance correspondante, que nous ratifions aujourd'hui et qui comporte quatorze articles seulement, a été prise en février 2017. De plus, l'ordonnance prévoyait la prise d'un décret d'application avant le 30 juin 2017 ; il n'a toujours pas été pris à ce jour Quelles qu'en soient les causes, comment admettre ces retards successifs ? Nos compatriotes d'outre-mer ne sont pas des citoyens de seconde zone : nous devons faire diligence pour adapter en temps utile le droit applicable localement. Sans doute devons-nous améliorer, madame la ministre, notre méthode pour légiférer pour les outre-mer : un rendez-vous annuel permettrait sans doute de mettre à niveau régulièrement, et sans retard excessif, les législations applicables localement, sans devoir s'en remettre trop souvent à des ordonnances. En première lecture, le Sénat a accepté de ratifier l'ordonnance, tout en y ajoutant trois dispositions : premièrement, par stricte analogie avec les règles déjà prévues par la loi pour l'Autorité nationale la fixation des délais de recours contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles et l'attribution à la cour d'appel de Paris de la compétence pour connaître de ces décisions deuxièmement, la détermination d'une base légale permettant à l'Autorité nationale de la concurrence et à l'Autorité polynésienne de la concurrence de coopérer volontairement dans le cadre d'enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles troisièmement, enfin, pour remédier à une malfaçon de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, le rétablissement, dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'obligation de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les déclarations d'intérêts et de patrimoine pour les membres, directeurs généraux et secrétaires généraux des autorités administratives indépendantes de régulation économique que peuvent créer non seulement la Polynésie française, mais également la Nouvelle-Calédonie, dans un strict parallélisme des formes et par stricte analogie, là encore, avec les règles applicables aux autorités administratives indépendantes nationales. L'Assemblée nationale a apporté à ces dispositions des modifications rédactionnelles ponctuelles, ne soulevant aucune difficulté, de sorte que la commission mixte paritaire les a approuvées. a approuvées. Elle a également ajouté deux dispositions supplémentaires, qui posent toutes les deux, à mon sens, des difficultés. D'une part, nos collègues députés ont fait mention des rapporteurs généraux des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, au titre des obligations déclaratives auprès de la HATVP, au motif que les deux seules autorités existantes -deux autorités de régulation de la concurrence -ont chacune un rapporteur général. Or, même si cette situation résulte de la même malfaçon de la loi Sapin 2, une telle obligation n'existe pas au niveau national pour le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, ce qui pose un problème au regard du principe d'égalité. avait bien identifié cette difficulté, mais nous avons considéré que celle-ci devait être résolue de façon globale, à l'occasion d'une prochaine révision de la loi relative à la transparence de la vie publique. La commission mixte paritaire s'est ralliée à la position du Sénat sur ce point. D'autre part, l'Assemblée nationale a introduit des dispositions visant à étendre à l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie certains pouvoirs d'enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles. Sur le fond, ce sont des dispositions analogues à celles qui sont prévues par l'ordonnance que nous ratifions concernant la Polynésie. La rédaction retenue me semble néanmoins perfectible, et je ne suis pas convaincue qu'elle fasse parfaitement la distinction entre ce qui relève de la compétence du législateur national, et que nous pouvons voter, et ce qui relève de celle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. De plus, elle omet la faculté de coopération avec l'Autorité nationale de la concurrence. Enfin, dans un texte propre à la Polynésie, introduire ces dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie, au dernier moment et sans expertise juridique suffisante, semble quelque peu cavalier. Néanmoins, dans un esprit de compromis et de responsabilité, au vu des besoins liés à la mise en place il y a quelques mois seulement de l'autorité calédonienne, mais aussi compte tenu du risque de caducité de l'ordonnance que nous devons ratifier, la commission mixte paritaire a accepté de conserver ces dispositions en l'état. Toutefois, je je prendrai l'initiative, dans les prochains mois, de proposer un texte afin de parfaire les dispositions concernant l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Sous le bénéfice de ces observations,

Monsieur le président, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, faire vivre la concurrence dans l'ensemble des territoires de la République, tel est le sens profond de ce projet de loi. C'est une exigence forte de nos concitoyens ultramarins, comme vous l'avez dit, madame la rapporteur. L'insularité, l'isolement géographique, ainsi que des structures économiques pas assez tournées vers la production locale, peuvent conduire à une déformation des prix au détriment du consommateur. C'est le thème de la « vie chère » qui demeure une préoccupation du quotidien, car c'est toujours le consommateur qui,, paie l'absence de concurrence et l'existence de situation de monopole. Si l'Autorité nationale de la concurrence est compétente dans les départements et régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, il n'en va pas de même pour les collectivités territoriales

Par une loi du pays du 23 février 2015, l'Assemblée de la Polynésie française a créé une autorité administrative indépendante, dotée de pouvoirs de sanction, l'Autorité polynésienne de la concurrence, l'APC. Cette loi est entrée en vigueur le 1 février 2016. L'ordonnance du 9 février 2017, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution et soumise aujourd'hui à votre ratification, a pour objet de prendre les mesures nécessaires afin que l'Autorité polynésienne de la concurrence puisse exercer pleinement ses fonctions et disposer enfin de moyens de contrôle coercitifs. Son décret d'application devrait, après bien des vicissitudes, être publié dans les prochaines semaines. Oui, madame la rapporteur, le temps a été trop long. Pour faire de ce texte de ratification une opportunité, le Sénat l'a enrichi-

répression des fraudes. Il a rétabli l'obligation de transmission de déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les membres des autorités administratives indépendantes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Dans le même esprit, l'Assemblée nationale a elle aussi apporté des compléments, pour étendre les obligations de déclaration auprès de la HATVP aux rapporteurs généraux des autorités polynésiennes et calédoniennes, dès lors que ceux-ci disposent de prérogatives significatives lors de l'instruction des affaires, et pour étendre certaines techniques d'enquête dont bénéficie l'Autorité nationale de la concurrence à l'Autorité calédonienne de la concurrence. L'accord obtenu en commission mixte paritaire permettra de ratifier l'ordonnance du 9 février 2017 dans les délais voulus : c'était essentiel. Je tiens à remercier tous les parlementaires qui se sont investis dans l'examen de ce sous un abord technique, touche à des préoccupations concrètes des habitants de Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Madame la rapporteur, je suis d'accord avec vous : il faut que les délais administratifs et législatifs soient plus respectueux

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, l'ordonnance du 9 février 2017 a été prise pour répondre aux attentes et aux besoins de l'Autorité polynésienne de la concurrence, créée en 2015, en la dotant des pouvoirs d'enquête nécessaires à la réalisation de ses missions. Si la Polynésie française a pu, par les lois du pays, créer une autorité administrative indépendante et adopter des réglementations de la concurrence et des pratiques commerciales, elle a dû, conformément à son statut, solliciter l'intervention de l'État pour que ce dispositif soit complété pour les matières relevant de la compétence de ce dernier en ce qui concerne le droit pénal, la procédure pénale et les voies de recours. Les mesures adoptées au travers de cette ordonnance reprennent largement les règles du livre IV du code de commerce, en les adaptant toutefois à la situation polynésienne. Conformément à l'article 74-1 de la Constitution, sur le fondement duquel elle a été prise, cette ordonnance doit nécessairement être ratifiée dans les dix-huit mois suivant Lors de son examen, en avril dernier, le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 9 février 2017 a reçu un large soutien de la part des sénateurs. Ainsi, l'article unique du projet de loi initial, valant ratification de l'ordonnance, a été adopté.

ont été adoptés en commission des lois, qui ont modifié le droit applicable à l'Autorité polynésienne de la concurrence. Le premier de ces amendements, devenu l'article 2 du projet de loi, tire les conséquences du retard du Gouvernement dans l'édiction du décret d'application de l'ordonnance en élevant au niveau législatif des dispositions relatives aux voies de recours. En outre, il organise la coopération en matière d'enquêtes de concurrence entre l'Autorité polynésienne de la concurrence et, au niveau national, l'Autorité de la concurrence ou les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Le second amendement, devenu l'article 3 du projet de loi, soumet les membres et les agents des grades les plus élevés des autorités de la concurrence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie à des obligations de déclaration d'intérêts et de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de façon à renforcer le contrôle déontologique dans ces institutions. Je me félicite que la commission mixte paritaire, qui fut conclusive, ait gardé l'ensemble des apports du Sénat. Elle a également conforté le travail de l'Assemblée nationale, qui a introduit l'article 4 portant extension de techniques d'enquête dont bénéficie l'Autorité nationale de la concurrence, pour lesquelles le législateur n'avait pas prévu d'application en Nouvelle-Calédonie depuis 2009. Cette extension, qui demeure dans le champ du projet de loi, puisqu'il s'agit de sanctionner des manquements au droit de la concurrence dans les deux territoires deux territoires ultramarins autonomes, concerne principalement les procédures en rapport avec les nouvelles technologies- saisies informatiques, identité d'emprunt. Madame la ministre, mes chers collègues, ce texte aux dispositions très techniques ne comporte aucune difficulté particulière et va dans le bon sens. En effet, il est nécessaire- c'était l'objet de l'ordonnance -de donner à ce territoire des instruments économiques et, à travers le code de commerce, les outils indispensables à la mise en oeuvre de la concurrence, à son contrôle et à son bon exercice. Aussi

Si l'image de l'outre-mer en métropole se résume parfois à une accumulation de clichés, le quotidien, pour les habitants, n'est pas toujours aussi paradisiaque. En effet, ceux-ci sont confrontés à l'éloignement géographique, à des difficultés économiques structurelles, comme le chômage et la vie chère, sans omettre les risques de catastrophe naturelle. Les cas de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ces lointains territoires du Pacifique sud, sont encore plus spécifiques. Les articles 74,75 et 76 de la Constitution leur confèrent une très large autonomie, y compris pour mettre en place des outils de développement et de régulation économique. Ainsi, la loi de 2012 relative à la régulation économique outre-mer ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, alors que, dans les départements ultramarins, elle a permis la mise en oeuvre du « bouclier qualité-prix et doté l'autorité de la concurrence de pouvoirs élargis, afin de lutter plus efficacement contre les oligopoles et la vie chère. C'est vrai ! Toutefois, l'État peut accompagner ces territoires autonomes, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait aujourd'hui par le biais du présent projet de loi. La Polynésie française est confrontée depuis plusieurs années à une crise du tourisme, à laquelle s'ajoutent des difficultés dans le secteur agricole, ainsi qu'un déficit en matière de développement industriel. Le niveau de vie y est plus faible qu'en métropole et le chômage, en particulier celui des jeunes, s'est fortement accru. Des caractéristiques plus structurelles, comme la part importante du secteur non marchand, le contrôle des prix et l'importation de la plupart des produits de consommation courante, viennent s'ajouter à ces faiblesses conjoncturelles. Pourtant, l'archipel est riche de nombreuses ressources paysagères, de sa faune et de sa flore uniques au monde, de la production locale de vanille, de coprah et de perles, et d'une zone économique exclusive aussi vaste que l'ensemble du continent européen. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, fait face à des problèmes comparables, même si son unité géographique-c'est le deuxième plus grand territoire ultramarin après la Guyane -, son moindre isolement- elle est située des côtes australiennes -et, surtout, la richesse de son sous-sol, en particulier ses gisements de nickel, en font un territoire bien doté. Il reste que, d'après l'Institut d'émission d'outre-mer, les prix en Nouvelle-Calédonie sont supérieurs de 33 % à ceux constatés en métropole, avec un écart record pour les produits alimentaires. Des coûts de production élevés, des marges confuses, la nécessité de stocker et le manque de concurrence entre les distributeurs expliquent ces prix élevés. À cela s'ajoutent les héritages de l'histoire et une situation politique dont nous connaissons la complexité. Le référendum prévu cet automne sera un rendez-vous crucial pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons voté il y a quelques mois la loi organique prévoyant les modalités de ce référendum. Nous savons que le Gouvernement est déterminé à ce que celui-ci se tienne dans les meilleures conditions possible pour l'avenir du territoire et de tous ses habitants. Si ce projet de loi n'a pas vocation à se situer au niveau de ces enjeux majeurs, il doit néanmoins apporter sa pierre à l'édifice juridique des deux territoires et contribuer ainsi à améliorer le fonctionnement des économies locales. L'ordonnance du 9 février 2017 renforce les pouvoirs d'enquête et de contrôle des agents de l'Autorité polynésienne de la concurrence, l'APC. Les apports du Sénat donnent à l'APC et à l'Autorité de la concurrence la possibilité de coopérer dans le cadre d'enquêtes. L'article 2 a également précisé les voies et délais de recours contre les décisions de l'APC, en consacrant naturellement la compétence de la cour d'appel de Paris en la matière. L'article 3, adopté dans la rédaction du Sénat, établit les obligations déclaratives des membres du collège de l'APC et de l'Autorité de concurrence de la Nouvelle-Calédonie à l'égard de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

concerne exclusivement la Nouvelle-Calédonie. Il permettra l'application de mesures de la loi Macron, de la loi de 2014 sur la consommation et de la loi de 2016 sur la lutte contre le terrorisme. Mon groupe apportera évidemment Mon groupe apportera évidemment son soutien à ces dispositions, qui relèvent d'une volonté de donner à ces territoires les moyens de leur développement. La vie chère est un mal endémique des territoires d'outre-mer, quoique nous connaissions aussi dans certains territoires métropolitains l'isolement géographique, l'enclavement même, et ses conséquences économiques et démographiques. Une autorité de la concurrence suffira-t-elle à résoudre ce problème ? Nous pensons que sa création est au moins de nature à y contribuer

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, les sénateurs du groupe La République En Marche ont accueilli avec grand intérêt ce projet de loi ratification de l'ordonnance étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence. L'extension du champ d'application territorial du droit de la concurrence à la Polynésie française nous apparaît comme une nécessité d'autant plus impérieuse, au regard de la bonne expression des mérites économiques, que ce territoire constitue un marché insulaire de modeste stature et se montre, en cela, peu enclin à endiguer la multiplication des positions monopolistiques abusives. La pertinence juridique de l'élaboration d'un droit de la concurrence applicable à la Polynésie française se passe de justifications supplémentaires, si bien que, dans un mouvement qui peut paraître anecdotique à certains, le Gouvernement nous enjoint de ratifier cette ordonnance. Il n'a pourtant échappé à personne qu'elle est prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution et que, par voie de conséquence, nous encourons le risque qu'elle soit frappée de caducité en l'absence de ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant sa publication. C'est toute la difficulté de l'exercice auquel nous sommes

Ce texte, rappelons-le, est issu d'une loi du pays du 23 février 2015, par l'entremise de laquelle l'Assemblée de la Polynésie française a institué une autorité administrative indépendante, l'Autorité polynésienne de la concurrence, dont les missions sont analogues à celles de l'Autorité de la concurrence nationale. Cette loi est entrée en vigueur le 1février 2016, mais l'application effective des mécanismes de régulation des relations commerciales en Polynésie française demeure limitée du fait de la répartition des domaines de compétence.

l'ordonnance soumise à notre ratification, élaborée à la demande de l'Assemblée de la Polynésie française, vise-t-elle à prendre les mesures nécessaires pour que l'Autorité polynésienne de la concurrence puisse exercer pleinement ses fonctions et soit pourvue d'instruments de contrôle coercitifs. examiné selon la procédure de législation en commission. Il a tiré les conséquences du retard gouvernemental dans l'édiction du décret d'application de l'ordonnance en élevant au niveau législatif des dispositions relatives aux voies de recours. En outre, il a organisé la coopération en matière d'enquêtes de concurrence entre l'Autorité polynésienne de la concurrence et, au niveau national, l'Autorité de la concurrence et les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il a rétabli l'obligation de transmission de déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les membres des autorités administratives indépendantes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette obligation n'existait plus à la suite d'une modification de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. À leur tour, les députés ont adopté le projet de loi qui leur était soumis. Voilà pour ces quelques éléments de cadrage. Mes chers collègues, hâtons-nous de réunir les conditions d'une concurrence économique saine dans nos territoires insulaires d'outre-mer. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons être assurés que c'est le consommateur qui, en bout de course, subira les conséquences de l'absence de réglementation en la matière. La Polynésie française est dans une dynamique positive en matière de concurrence, comme le montre la récente loi du pays du 14 mars 2018 interdisant les droits exclusifs d'importation et instituant une procédure de clémence minorant les sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre d'un opérateur économique en cas de dénonciation d'une pratique anticoncurrentielle à laquelle il a pris part. Nos régions ultramarines présentent des structures de marché distinctes de celles de la France hexagonale. L'établissement d'une autorité locale en matière de concurrence mérite d'être observé avec attention.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, si la loi polynésienne du 23 février 2015, entrée en vigueur le 1 février 2016, édictait un code de la concurrence et instituait une autorité polynésienne de la concurrence, calquée sur l'Autorité de la concurrence, il était nécessaire de la compléter pour les matières relevant de la compétence de l'État français. C'est l'objet de ce projet de loi, qui a été examiné selon la procédure de législation en commission. Comme le rappelait mon collègue Fabien Gay dans son explication de vote du 10 avril dernier, notre groupe politique a toujours considéré que la création des autorités administratives indépendantes s'inscrivait dans une forme de désengagement de l'État quant à la régulation des secteurs économiques les plus importants du pays

Cependant, en l'état du droit, ce projet de loi ne soulève, pour ainsi dire, pas de difficulté majeure. Nous concevons l'importance que revêt cette autorité de contrôle pour la Polynésie territoire insulaire où la conjonction d'une faible population- 280 000 habitantes et habitants -et d'un petit nombre d'acteurs économiques a tendance à favoriser la création de situations de monopole ou d'oligopole, d'ententes et de cartels qui pénalisent les consommatrices et consommateurs ultramarins. La commission des lois de l'Assemblée nationale a profité de ce véhicule législatif pour introduire un article concernant l'autorité néo-calédonienne Il s'agit d'actualiser et d'étendre les dispositions du code de commerce relatives aux pouvoirs d'enquête en matière de concurrence à la Nouvelle-Calédonie, afin que les agents de la direction des affaires économiques et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie disposent des mêmes pouvoirs que les agents assermentés en métropole pour la constatation des infractions à la réglementation économique. Cette autorité néo-calédonienne de la concurrence bénéficiera ainsi d'un cadre législatif lui permettant d'accomplir pleinement ses missions. Nous n'y sommes pas opposés. Finalement, compte tenu de l'accord trouvé en commission mixte paritaire, et respectueux de la volonté du législateur polynésien de se doter d'une autorité de la concurrence disposant des mêmes pouvoirs que l'autorité métropolitaine, les membres du groupe CRCE voteront en faveur de l'adoption

de Polynésie française, l'APC. Depuis sa création en 2015, l'APC a permis une évolution majeure dans l'environnement économique de l'archipel. Elle est le résultat de dix années de construction du droit de la concurrence polynésien dans un territoire complexe, sans doute unique, du fait de son isolement et de son éclatement territorial. Si l'APC dispose de pouvoirs similaires à ceux de l'Autorité de la concurrence nationale, aucune disposition n'était prévue concernant les pouvoirs d'enquête de ses agents ou les ou les voies de recours contre ses décisions. De telles dispositions relèvent en effet du domaine de compétences de l'État, et donc de notre Parlement. Ce projet de loi, qui prévoit la ratification de l'ordonnance, vise à remédier à cette situation et donnera à l'APC tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. Ainsi, ce texte complète les règles locales relatives à l'APC en matière de droit pénal, de procédure pénale, de procédure administrative contentieuse et d'organisation judiciaire. Il donne à l'APC une compétence juridictionnelle en matière d'indemnisation des préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles. Il attribue aux agents de l'APC un un pouvoir d'enquête qui leur permettra d'effectuer des contrôles dans les locaux à usage professionnel. Ces dispositions sont essentielles au regard de la lutte que la Polynésie française a engagée contre la vie chère et les situations de concentration de marchés. La Nouvelle-Calédonie, archipel voisin du Pacifique, s'est également dotée d'une autorité de la concurrence. La création de cette autorité, projet porté depuis 2009 par mon collègue député Philippe Gomès, a conclu un parcours long et tumultueux, qui n'a abouti que très récemment, puisque l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été officiellement installée le 2 novembre dernier. Il restait une dernière étape à franchir : étendre à la Nouvelle-Calédonie les nouveaux dispositifs d'enquête dont bénéficient aujourd'hui l'Autorité nationale de la concurrence et son homologue polynésienne.

Cet article permettra d'actualiser et d'étendre les dispositions du code de commerce en matière de concurrence à la Nouvelle-Calédonie. Les agents de la direction des affaires économiques et de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie pourront ainsi disposer des mêmes pouvoirs que les agents assermentés en métropole pour la constatation des infractions à la réglementation économique. est parvenue à un accord, notamment pour conserver l'article 4 dans le projet de loi ; je m'en félicite. Il aurait été dommageable de nous priver de ce véhicule législatif pour introduire une disposition aussi importante pour la Nouvelle-Calédonie. Je tiens à remercier mon collègue Philippe Bonnecarrère, membre de la commission mixte paritaire, pour son soutien. Aujourd'hui, grâce au texte que nous examinons, l'APC et l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie pourront se prononcer sur les questions de concurrence, étudier la compatibilité des règles de concurrence entre entreprises locales et, le cas échéant, sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit d'une avancée majeure pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste votera en faveur de l'adoption de ce texte important pour nos territoires dans le domaine de la lutte contre la vie chère et pour la construction d'un environnement économique sain et dynamique pour nos économies insulaires. La

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, je remplace mon collègue Jean-Pierre Sueur.

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.

le débat sur l'orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2017 La conférence des présidents a décidé de joindre la discussion générale de ce projet de loi au débat sur l'orientation des finances publiques. Dans le débat commun, la parole est à M. le ministre de l'action et des comptes publics. Merci pour ces

est moins élevé que ce qui était prévu en loi de finances initiale et inférieur à la prévision présentée par le Gouvernement au mois de décembre 2017. Ces résultats, rien ne les garantissait à notre arrivée aux responsabilités. En effet, nos objectifs en matière de finances publiques n'ont été atteints, et même dépassés, qu'à la faveur de la reprise en main des comptes publics par la nouvelle majorité. Je le souligne, les seules bonnes nouvelles fiscales n'auraient pas suffi à ramener le déficit

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons avoir collectivement conscience que ces bons résultats ne sont qu'une étape sur la voie de l'équilibre budgétaire. Je le rappelle, depuis plus de quarante ans, notre pays dépense bien plus qu'il ne produit.

Cette situation a une conséquence concrète, sur laquelle je souhaite attirer votre attention : malgré une nette réduction du déficit budgétaire, en 2017 le refinancement du stock de notre dette a nécessité l'émission de 185 milliards d'euros de titres sur les marchés financiers,

Enfin, la situation patrimoniale de l'État suffit à démontrer que le plus dur reste à faire. De ce point de vue, l'examen du projet de loi de règlement est l'occasion de rappeler les éléments de bilan de comptabilité de l'État. Premièrement, la situation nette de l'État est de moins 1 260 milliards d'euros. Nous savons que la comptabilité de l'État ne peut se comparer à celle des entreprises, ni d'ailleurs tout à fait à celle des collectivités, qui sont soumises à une règle d'or, mais cette situation signifie néanmoins que nous continuons à nous endetter, marginalement pour investir et majoritairement pour couvrir des dépenses courantes. Il ne s'agit donc pas d'un bon endettement. Deuxièmement, le résultat Deuxièmement, le résultat patrimonial, c'est-à-dire la différence entre les produits et les charges, est négatif à hauteur de 61 milliards d'euros. Troisièmement, les engagements hors bilan de l'État, c'est-à-dire ceux qu'il peut être amené à honorer, s'élèvent à 2 212 milliards d'euros. l'encours de la dette est de 1 710 milliards d'euros, en augmentation de près de 64 milliards d'euros par rapport à 2016. Ces chiffres ont tendance à se réduire, mais ils demeurent très importants.

Nous avons lancé de grands chantiers de transformation de notre économie, tout en nous attaquant résolument à la dette et au déficit. La France est enfin sortie de la procédure pour déficit public excessif, dans laquelle elle était engluée depuis dix ans. C'est une étape majeure dans le rétablissement de la confiance envers la France.

nécessaire pour reconquérir une crédibilité auprès de nos partenaires européens, qui attendent- et c'est bien normal -des preuves tangibles de nos efforts. Cette crédibilité retrouvée est précieuse pour nous permettre de jouer en Europe un rôle d'impulsion et d'orientation sur les enjeux majeurs. Sans respect de nos engagements, nous n'aurions certainement pas pu avancer sur la zone euro, ni aboutir à une feuille de route globale franco-allemande. Pour compléter la présentation faite par le ministre de l'action et des comptes publics de nos priorités en matière de finances publiques, je souhaite dire quelques mots des perspectives macroéconomiques de la France. Elles sont bonnes et doivent nous inciter à tenir le cap. L'économie française connaît une vraie dynamique de reprise depuis l'année dernière. La croissance a nettement accéléré, pour atteindre 2,3 % en 2017, alors qu'elle était proche de 1 % les années précédentes. Selon le scénario du programme de stabilité d'avril 2018, que nous reprenons, le dynamisme de l'activité se confirmerait, avec une croissance proche de 2 % en 2018 et en 2019. devrait être soutenue notamment par un environnement international qui reste porteur malgré les risques géopolitiques que nous connaissons tous, par l'investissement des entreprises et par des créations d'emplois toujours dynamiques dans le secteur marchand. Les données conjoncturelles publiées depuis l'élaboration du programme de stabilité font cependant état de signaux en léger repli. Cependant, elles n'appellent pas à ce stade de révision de notre scénario. Le ralentissement observé au premier trimestre est le contrecoup d'une année 2017 très dynamique. des enquêtes de conjoncture se stabilisent à des niveaux élevés et suggèrent que l'activité sera toujours soutenue en 2018. Nous verrons, lors de la préparation du projet de loi de finances, s'il y a lieu de réexaminer nos hypothèses de croissance au regard des nouvelles informations qui seront disponibles à cette date.

La situation des entreprises s'améliore, et leur investissement restera particulièrement dynamique, avec une croissance estimée à 4,4 %. La consommation des ménages bénéficiera au second semestre de baisses de prélèvements obligatoires importantes, la première tranche de la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales ou la revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adultes handicapés. Ces mesures viendront soutenir la consommation des ménages en fin d'année. Le pouvoir d'achat devrait donc continuer à croître en 2018.

aujourd'hui, malgré les progrès déjà réalisés, notre économie souffre de plusieurs maux, et nous avons encore de larges marges de progrès. C'est le cas en matière de compétitivité : un regard sur nos performances à l'export suffit à s'en persuader. C'est vrai aussi en matière de productivité : notre économie doit moderniser ses capacités productives, accroître son effort en matière d'investissement et d'innovation. En matière d'emploi, il est grand temps que le chômage de masse, qui touche encore près de 9 % de nos concitoyens, reflue vraiment. Notre réponse, c'est une vraie transformation structurelle de notre économie, en trois volets. Le premier consiste à libérer le plein potentiel de notre économie pour déverrouiller la croissance et l'emploi. Pour cela, nous avons entamé une profonde réforme du marché du travail, notre philosophie étant d'accorder une place centrale à la négociation collective et de permettre aux entreprises d'embaucher en toute sécurité. Cette souplesse va de pair avec la sécurisation des parcours professionnels, les réformes de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Par ailleurs, nous favorisons l'investissement, car c'est en investissant que nous voulons restaurer notre compétitivité. travers du budget pour 2018, nous avons engagé une vraie révolution fiscale. L'objectif est d'alléger et de simplifier la fiscalité sur le capital, afin que nos entreprises se financent mieux et plus facilement, et soient donc plus solides.

Le deuxième volet de cette grande transformation est celui de la préparation de l'avenir. Dans chaque secteur-clé de l'économie, nous entendons combiner réformes structurelles et politique ambitieuse d'investissement. Nous créons un fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation de rupture et le développement de notre stratégie pour l'intelligence artificielle. Nous investissons massivement dans l'éducation, l'apprentissage et la formation professionnelle.

loi PACTE, nous allons aussi poser les fondements d'une confiance retrouvée avec l'entreprise. Nous encourageons le développement de l'intéressement et de la participation, pour permettre aux salariés d'être mieux récompensés pour la réussite de leur entreprise. Nous sommes convaincus que notre capacité à réformer repose sur notre capacité à restaurer l'équilibre de nos finances publiques. Dans un pays où la dépense publique représente 56 % de la richesse nationale, la transformation de notre modèle économique et social passe nécessairement par une transformation de nos services publics. améliorer l'efficience de nos services publics et ainsi mieux maîtriser les dépenses ; baisser les impôts pour redonner des marges de manoeuvre aux entreprises et aux ménages ; réduire sensiblement la dette pour réduire notre vulnérabilité en cas de crise et les charges pesant sur les générations futures. En 2017, le déficit s'est établi à 2,6 % du PIB. En 2018, il sera de 2,3 %. Nous diminuerons les prélèvements obligatoires et la dépense publique, une dépense publique que l'on a trop souvent utilisée comme une solution miracle à tous les problèmes économiques et sociaux, sans traiter les causes profondes. Enfin, nous réduirons la dette. C'est indispensable pour faire baisser le service de la dette, qui est de l'argent public jeté par les fenêtres, et pour nous protéger contre une remontée des taux. Une hausse d'un point des taux d'intérêt aujourd'hui entraînerait 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dès cette année, et près de 16 milliards d'euros

L'in constate aussi des trajectoires contrastées entre les sous-secteurs de l'administration publique. En effet, si les administrations publiques locales et les administrations sociales enregistrent un solde positif, l'État reste très fortement déficitaire, à hauteur de près de 60 milliards d'euros.

mes chers collègues, en 2017, pour la première fois depuis l'éclatement de la crise financière, les comptes des administrations de sécurité sociale, les ASSO, sont revenus à l'équilibre,

elle est appelée à disparaître le jour où elle aura achevé sa mission. Or, si l'on s'intéresse aux résultats des autres ASSO- les ASSO pérennes, en quelque sorte

En deuxième lieu, monsieur le ministre, l'embellie des comptes des ASSO est largement due à la forte augmentation des recettes des différentes administrations de sécurité sociale. Poussées par la bonne conjoncture économique et par l'augmentation, inattendue par son ampleur,

ce constat ne se vérifie pas au niveau des sous-objectifs, la sous-exécution des établissements de santé compensant, en quelque sorte, la surexécution des soins de ville. Selon l'avis du comité d'alerte sur le respect de l'ONDAM, cette situation aurait encore empiré en 2018. Au vu de la situation des hôpitaux, une telle trajectoire n'est plus supportable. Nous attendons donc avec impatience les annonces du Gouvernement en matière d'organisation de notre système de santé. Après ce rapide coup d'oeil dans le rétroviseur, qu'en est-il de 2018 et des années suivantes ? annonce une « amélioration durable de l'équilibre des comptes sociaux ». Plus précisément, l'excédent des ASSO connaîtrait une nouvelle amélioration dès cette année 2018, pour atteindre 0,7 point de PIB. De fait, la commission des comptes de la sécurité sociale prévoit un quasi-retour à l'équilibre de l'ensemble régime général-FSV, avec un déficit ramené à 300 millions d'euros seulement. Par la suite, on le sait, un excédent de 0,8 point de PIB est prévu jusqu'en 2022, avec un plafonnement de ce solde par l'État. Nous serions donc enfin revenus de façon robuste et durable à l'équilibre des comptes sociaux. Pourtant, monsieur le ministre, j'ai indiqué à la commission des affaires sociales que, à ce stade, cet équilibre demeure instable, en raison en raison notamment des quelques incertitudes d'ordre juridique qui planent sur le solde de 2018. Je pense par exemple à la question de la compensation à la sécurité sociale du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, le CITS. L'enjeu, de l'ordre de 600 millions d'euros, est de nature à empêcher les comptes du régime général et du FSV de tutoyer l'équilibre dès cette année. Mes interrogations sont plus fondamentales et de plusieurs ordres. Elles concernent, tout d'abord, la croissance. Madame la secrétaire d'État, vous avez parlé des prévisions Plus encore que ceux de l'État, les comptes des ASSO sont sensibles à la conjoncture : en recettes, à cause d'une forte corrélation de leur évolution avec celle de la masse salariale, et parfois en dépenses, notamment dans le cas emblématique de l'assurance chômage. Pour 2018, nous l'avons vu, les prévisions actualisées anticipent un ralentissement de la croissance à 1,7 %, selon l'INSEE, après les 2,3 % de 2017, un chiffre donc des 2 % qui figurent dans le rapport du Gouvernement. Surtout, pour la suite, le Gouvernement prévoit un taux de croissance de 1,9 % en 2019, puis de 1,7 % entre 2020 et 2022. Comme le relève la Cour des comptes, ce scénario fait le pari d'une croissance réelle supérieure à la croissance potentielle

Le taux de croissance en volume des dépenses des ASSO figurant dans la loi de programmation des finances publiques est compris, selon les années, entre 0,1 % et 0,9 %. Or les quelques éléments connus

Il faudra donner au coup de frein sérieux aux autres dépenses pour que la trajectoire soit tenue, mais les économies envisagées ne sont pas documentées pour le moment

ou encore des mesures relatives à l'indemnisation du chômage des démissionnaires et des indépendants. J'ajouterai même qu'il sera difficile de réaliser une grande réforme des retraites, avec un objectif de justice sociale, à coûts constants.

sur la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Nous l'attendons évidemment avec impatience ... On le voit, il y a de quoi remettre en cause la trajectoire financière apparemment favorable des ASSO pour les années qui viennent.

Si, en soi, le retour à l'équilibre des comptes sociaux en 2017 est une bonne nouvelle, de réels facteurs d'instabilité pèsent encore sur la trajectoire financière des ASSO. Certes, il n'est pas illégitime de repenser

cette révision doit se faire dans le respect de principes simples, que je souhaite rappeler. Tout d'abord, tant que subsistera une dette de la sécurité sociale, qu'elle soit portée par l'ACOSS, l'Agence centrale des

la CSG, pour les régimes universels- maladie, famille et peut-être, demain, dépendance -et des compensations simples, par exemple crédits budgétaires ou TVA, pour la compensation du financement de politiques de l'État.

nous avons toujours plaisir à vous retrouver ! Le plaisir est partagé ! Assurance en toutes circonstances, affirmations toujours discutables, morgue parfois, provocation toujours Nous examinons donc cet après-midi le projet de loi de règlement, couplé au débat sur l'orientation des finances publiques pour 2019. Concernant le projet de loi de règlement du budget de l'année 2017, nous pouvons en faire deux lectures, qui ont chacune du sens. S'il s'agit de savoir si l'exécution des crédits est en adéquation avec la loi de finances pour 2017, corrigée des décrets d'avance et modifications apportées en loi de finances rectificative, notamment du fait de l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale en cours d'exercice, ce projet de loi est conforme. Il fait apparaître que l'amélioration de la croissance et un retour à un taux supérieur à 2 %, résultat de la politique conduite par vos prédécesseurs, permettaient en toute hypothèse le retour du déficit public en deçà de 3 les mesures d'économies prises, selon le rapport de notre excellent rapporteur général de la commission des finances, portant sur 1,5 milliard d'euros, soit moins de 0,1 % du PIB. Autrement dit, sans les mesures que vous avez prises en toute hâte, le déficit aurait été ramené à 2,7 %, au lieu de 2,6 % : telle est la simple réalité des choses Au passage, notons que 2,7 %, c'était l'objectif précis de l'ancienne équipe, résultat- reconnaissons-le -qui ne pouvait être atteint qu'avec une croissance plus forte que celle projetée en loi de finances initiale. définitive, vous avez préféré instrumentaliser un document de la Cour des comptes pour prendre des mesures qui se sont révélées limitées dans leurs effets et inutilement brutales dans leur application, que ce soit en matière de contrats aidés ou d'aides

S'agissant des dépenses de l'État, la Cour estime à 1,5 milliard d'euros les tensions liées à des " sous-budgétisations ". Nous regrettons vivement le choix de ce terme, qui laisse à penser que le Gouvernement a volontairement minoré certaines dotations en loi de finances. Si des tensions peuvent exister, elles sont le fruit des aléas naturels qui apparaissent en gestion » ... C'est beau comme l'antique ! C'est l'ancien Ainsi donc, la Cour des comptes chiffre à 1,5 milliard d'euros les sous-budgétisations de votre budget pour 2018 ... Je comprends que vous vous en émouviez L'année dernière, j'indiquais que le rapport de la Cour des comptes portant sur l'exécution du budget pour 2018 serait sans doute moins commenté. Nous n'avons pas eu longtemps à attendre pour que, à votre tour, vous vous agaciez. Mais rassurez-vous : sous-budgétisation aujourd'hui, éléments d'insincérité demain ... Vous n'en avez pas fini avec les appréciations de la Cour des comptes ; comptez sur nous pour vous en rappeler régulièrement les termes

des éléments essentiels d'information, alors que ce débat est censé préfigurer les orientations du projet de loi de finances à venir. Je constate d'abord que le « tiré à part » qui retrace l'évolution future des missions budgétaires ne nous a été remis qu'hier, en fin d'après-midi. En outre, ce document, pour une fois, ne comporte pas d'indications sur l'évolution des effectifs par mission. Cette pratique, qui n'est hélas pas nouvelle, est d'autant plus surprenante que, parallèlement, vous affirmez -sans rire -vouloir renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement ! Lors de la présentation du programme de stabilité pour la période 2018-2022, vous n'hésitiez pas à considérer, contre toute analyse sérieuse, que quelques mois d'action gouvernementale étaient à l'origine d'une croissance de 2,2 % en 2017 2017, tous les organismes sérieux mettent ces résultats au crédit du gouvernement Hollande : c'est ainsi ! En 2018, les mesures prises à la par votre gouvernement et le choc de confiance que vous revendiquiez produisent leurs premiers effets. Et quels effets ! Croissance trimestrielle retombée à 0,2

Ces éléments auraient sans doute mérité d'être mieux mis en lumière. D'autres sujets sont discrètement traités : l'abandon de la taxe d'habitation se traduit par un appel supplémentaire à l'emprunt ; la reprise de la la reprise de la dette de la SNCF donne lieu à un propos nébuleux à ce stade ; la baisse annoncée de la dépense publique n'est toujours pas sérieusement documentée ; les travaux d'Action publique 2022 n'ont toujours donné lieu à aucune communication, ni sur les propositions faites par ce par ce fameux comité ni sur celles retenues par le Gouvernement. Votre rapport fait également l'impasse sur la fin de l'imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelée. Au-delà de la logique politique qui sous-tend cette décision du Président de la République, à laquelle nous nous opposons- c'est un débat que nous aurons lors de l'examen du projet de loi de finances -, quel en sera exactement l'impact comptable ? C'est une question intéressante à soulever, me semble-t-il, dans le cadre d'un débat sur l'orientation des finances publiques. Or le manque à gagner, pour les finances de l'État, a fait l'objet d'évaluations très diverses : 803 millions d'euros selon le Conseil des prélèvements obligatoires, mais 2,5 milliards d'euros de créances potentielles selon le Gouvernement. Puis, dernièrement, Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale, a déclaré devant les députés que « le stock d'impôt sur les plus-values latentes au titre de l'était de 6 milliards d'euros », mais que son rendement réel est de 140 millions d'euros depuis 2012 Ces estimations divergentes nous laissent particulièrement perplexes, pour ne pas dire pantois ! Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, quel sera le coût réel de la suppression de l'pour le budget de l'État ? Le débat sur l'orientation des finances publiques est aussi le moment de discuter de la trajectoire et de l'équilibre des comptes sociaux. Sur ce point encore, nous sommes dans le flou. Le 20 mai dernier, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a déclaré que, « à partir du moment où nous réussissons à créer des [postes] dans le secteur privé [ ...] il peut être légitime de réduire la politique sociale sur l'emploi ». Quelques jours plus tard, vous avez pour votre part estimé, monsieur le ministre, qu'il ne fallait « pas toucher aux prestations sociales individualisées Puis la ministre de la santé, Agnès Buzyn, a assuré devant l'Assemblée nationale qu'il n'y aurait « pas de remise en cause des aides sociales ». Enfin, vous avez déclaré, le 29 mai, qu'« il y avait trop d'aides sociales en France » et que le système social devait être revu, mais « sans jamais diminuer les prestations individuelles des gens

presse, décidément toujours mieux informée que le Parlement, s'est d'ailleurs fait l'écho de plusieurs pistes d'économies. Là encore, ces informations ne sont pas évoquées dans le document que vous nous avez remis. Sans doute s'agit-il d'un oubli ... De tout cela, que devons-nous retenir, monsieur le ministre ? Ce qui apparaît clairement aux yeux de tous, c'est qu'après vous être attribué indûment les résultats de vos prédécesseurs, vos premiers résultats réels sont plus que décevants, et que vous hésitez tellement sur vos propositions budgétaires futures que vous avez préféré vider de son contenu ce débat sur l'orientation des finances publiques. Transparence, disiez-vous ? Bravo ! La parole

Merci

D'espoir d'abord, car la croissance a été robuste en 2017 : 2,2 %, c'est un rythme que notre économie n'avait plus connu depuis la crise. Cette loi de règlement est donc aussi une loi de rémission pour l'économie française. Elle entérine le retour de la France sur un sentier de croissance stable, un peu au-delà de sa croissance potentielle. Cette croissance permet au pays d'afficher un déficit public nominal de 2,6 % du PIB à l'issue de l'exercice 2017 et de sortir de la procédure pour déficit excessif. J'entends, bien sûr, la réserve : c'est grâce au dynamisme des recettes. C'est un fait, mais cela n'occulte pas le fait que la France retrouve peu à peu sa crédibilité en Europe, une crédibilité qui lui sera nécessaire pour prétendre réformer la zone euro. les comptes des administrations de sécurité sociale retrouvent en 2017 un solde positif, en attendant les excédents du régime général de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse, prévus dès 2019. Mes chers collègues, cela n'était plus arrivé depuis 2002

l'inquiétude des collectivités, qui doivent faire face à la réforme de la taxe d'habitation et aux incertitudes concernant leur autonomie financière. Je pense particulièrement aux départements, dont la situation est critique face à des dépenses sociales dont ils n'ont pas la maîtrise et qui sont en croissance permanente.

Après l'espoir, les craintes, puisque Spinoza disait qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Allons bon ! La crainte principale tient à l'incapacité structurelle de notre pays à réduire sa dépense publique. Nous n'y arrivons pas Nous avons beau faire des revues de dépenses, des RGPP ou des MAP, créer des directions interministérielles de la transformation publique ou des secrétariats généraux à la modernisation de l'action publique, et commander des rapports à de hauts fonctionnaires, force est de constater que nous n'y arrivons pas.

Il faudra un grand volontarisme politique pour porter cette question ; nous ne pourrons pas toujours compter de bonnes nouvelles en recettes. Notre position, ici, au Sénat, est très confortable, et j'ai l'habitude de dire « Que ferions-nous si nous étions aux affaires ? Derrière chaque niche, il y a un chien ; derrière chaque poste, il y a un syndicat ; Eh oui ... ... derrière chaque politique publique, il y a un électeur. Il vous faudra donc faire preuve de courage politique pour rendre les arbitrages nécessaires. C'est ce que commande l'intérêt supérieur de la Nation. Je sais que ce n'est pas une tâche aisée. En effet, quelle est la situation aujourd'hui ? Notre dette a continué de croître en 2017, notre pays est le seul grand État de la zone euro à ne pas avoir débuté son désendettement- M. le rapporteur général de la commission des finances le rappelle régulièrement. L'Allemagne, les Pays-Bas et même le Portugal se désendettent autant en un an que ce que nous ferons en cinq ans, et nous avons un écart d'endettement de plus de 30 points de PIB avec l'Allemagne. Cette situation est critique pour au moins trois raisons. La première est que notre marge de manoeuvre budgétaire est quasi nulle pour faire face à une nouvelle crise ; or les nuages s'amoncellent sur l'économie et sur les bourses mondiales. La deuxième est que nous risquons de ne plus avoir les moyens de nos ambitions politiques, et nous mettons en péril notre souveraineté et notre influence dans le monde.

nous devons nous tourner vers l'avenir. Ce débat d'orientation budgétaire est donc celui de l'espoir et des craintes. Il ne tient qu'à vous, monsieur le ministre, comme Spinoza vous y invite, d'alimenter nos espoirs et d'apaiser nos craintes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, au travers de ce projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2017, le Gouvernement constate un déficit budgétaire de 67,7 milliards d'euros,

Comme je l'avais indiqué lors des débats sur la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, ce résultat s'inscrit dans une trajectoire qui semble crédible, malgré les incertitudes macroéconomiques, qui rendent par essence toute prévision difficile.

Le dérapage des dépenses publiques, qui aurait pu être plus marqué sans un effort de rigueur du nouveau gouvernement, est bien à imputer à l'ancienne majorité.

l'embellie en matière de recettes est la conjonction de mesures antérieures à 2017 et d'un effet d'accélération lié au dynamisme et au programme de réforme du président élu en mai 2017 et de la nouvelle majorité. Avec un déficit des administrations publiques ramené à 2,6 % du PIB en 2017, plus faible que les prévisions les plus optimistes, la France respecte pour la première fois depuis une décennie ses engagements européens, ce qui lui permet de sortir de la procédure de déficit public excessif. Ce bon résultat découle d'une croissance d'un niveau inattendu l'an dernier, qui tient pour partie à un effet de rattrapage, constaté également chez nos voisins européens, et pour partie au choc de confiance suscité par l'arrivée d'un nouvel exécutif, porteur d'une nouvelle ambition pour la France du point de vue des réformes, du dynamisme et du rayonnement. Enfin, il faut reconnaître que l'instauration de la contribution exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros fondée sur l'impôt sur les sociétés a permis de neutraliser l'annulation de la taxe de 3 % sur les dividendes. Sans cette mesure, le résultat budgétaire aurait été sensiblement différent.

Compte tenu de ces différents éléments, on voit bien que le principal enjeu pour l'exercice budgétaire présent et les suivants sera la maîtrise des dépenses. Contrairement à ce que l'on entend parfois, l'appareil administratif français n'est pas « à l'os trois agences au début des années 2000, en compte aujourd'hui plus d'une soixantaine. Le maintien de technostructures de toutes natures, souvent inutiles, et de doublons dans certains territoires suscite des interrogations quant à la répartition et à l'efficacité de la gestion de certaines compétences publiques.

Aussi le Gouvernement est-il très attendu sur ces différents points. Les mesures annoncées de réorganisation territoriale et de contraction d'effectifs au sein du ministère des finances, à condition qu'elles soient menées avec discernement, vont, me semble-t-il, dans le bon sens, et la méthode doit pouvoir être appliquée à d'autres ministères, qui intègrent des services parfois totalement étrangers à leurs missions régaliennes. Dans son rapport de l'an dernier, la Cour des comptes recommandait déjà une baisse de la dépense publique plus sélective, plus structurelle et accompagnée de véritables programmes d'investissement. Vu les documents qui nous ont été fournis, force est de constater les disparités entre les différentes catégories d'administrations publiques. Il en ressort que ce sont les administrations centrales, donc l'État et ses nombreuses excroissances, qui sont responsables de la plus grande part du déficit, alors que les collectivités locales sont à l'équilibre- elles ont d'ailleurs l'obligation d'appliquer la règle d'or budgétaire, qui leur interdit d'adopter un budget en déficit. en déficit. Les administrations de sécurité sociale connaissent, quant à elles, un léger excédent, même si l'impact social, en particulier à l'hôpital, doit être suivi de près. le projet de réforme du calendrier budgétaire présenté dans le cadre de projet de réforme institutionnelle, on ne peut que souscrire à la volonté de renforcer les capacités de contrôle et d'évaluation du Parlement en la matière, comptes sociaux Un rééquilibrage entre la loi de finances initiale et la loi de règlement, en faveur de cette dernière, semble souhaitable. L'objectif central du Gouvernement doit demeurer, en la matière, la préservation du Parlement comme lieu privilégié de proposition, d'examen, de débat, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Anticipant l'examen du projet de loi de finances pour 2019, je n'évoquerai que la grande novation qu'est le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Je dis « novation », et non « innovation », parce que cette imposition est pratiquée dans de nombreux pays et que les deux autres principales ressources fiscales, la TVA et l'IS, sont déjà collectées par les entreprises. Absolument ! Cette réforme, longtemps repoussée, décidée par le précédent gouvernement, reportée d'un an puis reprise par ce gouvernement, est désormais actée. Si les attentes concernant sa mise en oeuvre technique sont fortes, la décision du Gouvernement de reporter à nouveau son entrée en vigueur pour les salariés de particuliers peut être interprétée comme une preuve de pragmatisme et de souplesse- si l'on voit les choses de manière optimiste comme avec la mise en place de tout dispositif nouveau, à quelques difficultés et ajustements, les inconvénients et les coûts ponctuels ou récurrents de cette réforme semblent avoir été très largement surestimés par certains. En conclusion, si je comprends bien les contraintes et les objectifs macroéconomiques du Gouvernement, j'invite ce dernier à se montrer davantage à l'écoute des territoires ruraux, des villes petites et moyennes, des quartiers périurbains, c'est-à-dire de toute la France dite « périphérique des préoccupations de leurs élus et de leurs habitants. Veuillez conclure, mon cher collègue. Nous prenons bonne note de l'intention du Président de la République, annoncée lors du Congrès à Versailles, d'un rééquilibrage des territoires et de la mise en oeuvre d'un principe de différenciation.

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs généraux, chers collègues, nous sommes aujourd'hui à un moment important du calendrier budgétaire. Il s'agit d'abord de voter la loi de règlement de l'année dernière, en mettant en perspective l'action en matière budgétaire, de faire le point sur l'exécution de la loi de finances que nous avons adoptée, enfin de définir les perspectives pour l'année à venir. L'exercice 2017 a été une année de remise en ordre dans les finances publiques. Il a fallu faire face à l'impasse de financement de 8 milliards d'euros pointée par la Cour des comptes dans son audit de juin 2017 et à l'annulation de la taxe de 3 % sur les dividendes. Grâce à un effort de 5 milliards d'euros en recettes et de 5 milliards d'euros en dépenses, la sortie de la procédure pour déficit excessif a été actée.

Si la fin de la procédure pour déficit excessif pour la France doit être appréciée, la dette publique est en revanche en légère progression : elle s'élève à 96,8 % du PIB en 2017, contre 96,6 % en 2016, soit une hausse de 0,2 point du PIB. Un niveau inédit, qui a contraint le Gouvernement a entamé, dès le budget pour 2018, une démarche visant à réduire le poids des dépenses publiques, en passant d'une gestion budgétaire heurtée- mise en réserve, décrets d'avance, annulations de crédits -à une gestion plus respectueuse de l'autorisation parlementaire, en réduisant de 8 % à 3 % la mise en réserve des crédits. Résultat, l'évolution de la dépense publique passera de 1,5 % du PIB en 2017 à environ 0,7 % en 2018. Il s'agit de l'évolution la plus contenue depuis 2011, au lendemain du plan de relance de 2010.

pays. Nous devrons collectivement être attentifs à cet objectif. C'est pour cela que la loi de programmation des finances publiques adoptée par le Parlement définit une trajectoire sincère et ambitieuse pour nos comptes publics. Elle traduit les engagements pris par le Président de la République durant la campagne électorale et réaffirmés depuis lors avec constance. Aussi le cap du sérieux budgétaire sera-t-il maintenu en

Cet allégement fiscal pour tous les Français, je vous le rappelle, se traduira par une baisse de 5 milliards d'euros d'impôts en 2018, de 9 milliards en 2019 et de 7 milliards en 2020. C'est un geste sans précédent pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes et pour les entreprises. Retrouver l'équilibre budgétaire et faire baisser la dette nationale, oui, mais tout en favorisant la croissance de long terne et la confiance de nos concitoyens, de nos entreprises et de nos partenaires à l'étranger.

effet dans cette enveloppe qu'ont été puisés jusqu'à maintenant tous les moyens pour faire face aux difficultés exceptionnelles- crise en Guyane et à Mayotte, cyclones Maria et Irma aux Antilles. En d'autres termes,

Il s'agit seulement de la moyenne obtenue, lors des épreuves du baccalauréat, par une jeune fille de dix-huit ans, scolarisée en Polynésie, et qui, par la grâce de Parcoursup, se retrouve aujourd'hui sur liste d'attente dans un lycée métropolitain pour intégrer une classe préparatoire de mathématiques, faute de proposition en concordance avec ses attentes.

traduit le bilan d'une année de transition entre une majorité libérale qui s'est éloignée du social et une majorité qui organise le coup d'État de la finance contre le social et contre la démocratie. Il nous faut bien en dresser le bilan. Coup de tabac sur le prix de l'essence et du gaz, désencadrement des loyers, explosion de la précarité au travail avec le développement des plateformes et les effets conjugués des lois El Khomri et des ordonnances Pénicaud. 29 % des contrats de travail signés depuis le début de l'année sont des contrats d'un jour, monsieur le ministre- un seul jour ! Pour faire Pour faire bonne mesure, les prix recommencent à augmenter, pendant que l'on gèle le point d'indice, que l'on bride la progression du SMIC, que l'on maintient la rémunération du livret A sous l'évolution de l'indice des prix, que l'on compresse la dépense publique, que l'on diminue les APL et que l'on ponctionne les retraités avec la CSG N'allons pas chercher ailleurs les motifs de l'insatisfaction relative de l'opinion publique devant la politique menée ... Si l'on considère le rapport de la Cour des comptes ou que l'on se souvient des déclarations du gouverneur de la Banque de France, on comprend vite qu'il ne suffira pas d'habiller ce capitalisme de vertus pour qu'il porte enfin les remèdes opératoires nécessaires à sortir la France de l'ornière de la crise. On nous dit que les déficits ne baisseraient pas assez vite, mais est-il est-il seulement venu à l'idée des brillants experts en politique économique et budgétaire que ce sont précisément les recettes qu'ils appliquent qui repoussent sans cesse le moment où nous retrouverons l'équilibre ? Vous avez voulu alléger les cotisations sociales sur les bas salaires ? Fort bien, l'objectif est atteint ! Nous dépensons plus ou moins 30 milliards d'euros par an à entretenir ce que j'appelle le « tiers secteur » de la population active, active, ces millions de salariés à temps partiel, journaliers et autres, qui seront bientôt dépossédés de droits syndicaux, de droit à la formation et à la promotion sociale. Et nous avons dépensé, depuis 2012, quelque 60 milliards d'euros de CICE pour restaurer les marges des entreprises- objectif atteint, je vous rassure -, mais sans relance de l'investissement ni création massive d'emplois, sinon d'emplois précaires. Il est temps de dire « stop », d'autant que la Banque de France nous indique que la dette privée,

sur l'encombrement aux urgences, sur la mise en question des prestations familiales ou sur le gel des retraites et sur la hausse des prix ? Quand cessera ce procès instruit à l'encontre de la sécurité sociale, accusée d'être une charge pour la société, alors qu'elle constitue, au contraire, l'un des atouts du redressement économique et social du pays ? Il est temps de mettre de côté le traité budgétaire et la loi de programmation des finances publiques ; il est temps de stopper cette confusion que l'on entend régulièrement, y compris ici, entre économie et financiarisation ; il est urgent de remettre au coeur du débat la question de la croissance et de son contenu, question très bien illustrée dans le document. Selon nous, la croissance n'a pas de sens lorsque sa visée se réduit à gonfler les actifs du CAC 40 ; elle a en revanche du sens quand elle fait de l'emploi sa priorité. pas l'emploi déqualifié, maintenu sous perfusion par injection d'argent public à fonds perdu depuis trente ans, au grand bonheur des détenteurs de dette publique et de chefs d'entreprise à courte vue, non, l'emploi qualifié, reconnu par une véritable qualification et un salaire à la hauteur des besoins du temps ! Nous avons, mes chers collègues, 6 millions de salariés dans le halo du chômage et de la précarité, ayant une vie en pointillé, faite de difficultés quotidiennes, et nous avons entre 800 000 et 900 000 jeunes partis pour l'étranger pour travailler, faute de trouver en France l'emploi qu'ils méritent au regard de leur formation initiale. Ce sont l'absence totale d'audace d'une partie du patronat,

continue, depuis sa privatisation, à rechercher les investissements à retour rapide, et nous avons les vecteurs de la crise en cours et des catastrophes à venir. Il est temps que la puissance publique prenne la main dans cette affaire, ne serait-ce que pour donner une impulsion à l'activité. Les taux d'intérêt demeurent faibles ; mais qu'attend la France qu'attend la France pour négocier, au plus haut niveau européen, les enveloppes financières nécessaires à la mise en oeuvre de projets fondamentaux pour l'aménagement du territoire de notre pays comme de celui de l'Europe de demain ?

au titre de la suppression de la taxe d'habitation. Ce serait un message de confiance envoyé par le Gouvernement à l'ensemble des collectivités territoriales. Nous avons mieux à faire avec l'encours du livret A

vous avez un temps d'avance, oui, un temps d'avance sur le débat de la réforme institutionnelle, qui va concerner les lois de finances. Pourquoi ? Loi de programmation des finances publiques, programme de stabilité, débat d'orientation des finances publiques, loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale ; il y en a trop, et vous venez de montrer, au travers du document que vous avez livré, que le débat d'orientation des finances publiques ne servait plus à rien. Ce document est indigent : peu chiffré, pas de plafond d'emplois, pas de trajectoire crédible, non documenté. Pas d'insincérité non plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce document

C'est pour cela que je le précise. Venons-en à la loi de règlement. Je suis très heureux, que nous soyons sortis de la procédure de déficit excessif. Enfin ! La France était quasiment le dernier pays d'Europe dans cette situation. Ce n'est quand même pas une grande gloire, mais ça nous permettra de continuer à donner des leçons au reste du monde.

peu fortement ; l'improvisation de la situation a fait que vous avez dû mener une politique de incompréhensible sur les contrats aidés et faire des annonces difficiles sur les aides au logement ; tout cela a largement perturbé votre message. donc surtout grâce à la croissance et aux recettes que nous sommes sortis de ce déficit excessif, mais, je le répète, je suis content qu'il y ait de la croissance. Néanmoins, je n'ai pas toujours confiance dans la météo pour avoir chaud.

de la Banque de France, qui a écrit au Président de la République au mois de juin dernier, il y a, dans la sphère sociale, des économies à faire partout- pas forcément sur les prestations, mais dans la gestion

des sondages du Président de la République. Ça l'est davantage si c'est aux dépens des Français. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chaque année, nous dénonçons le peu de temps dont nous disposons pour examiner le projet de loi de règlement.

Elle a notamment permis de réduire le déficit public de la France et de repasser en dessous de la fameuse barre des 3 %, sortant ainsi de neuf années de procédure pour déficit excessif. Le Gouvernement tend à s'attribuer le bénéfice de cette amélioration du déficit. À dire vrai, la réalité est un peu différente, car cette amélioration s'explique, pour l'essentiel,

par cinq raisons : une hausse de 1 % du taux de croissance du PIB ; une augmentation de 1 point de l'investissement, grâce notamment à la hausse de 5 points des dépenses d'investissement des collectivités territoriales territoriales ; un excédent budgétaire de 5 milliards d'euros des administrations de sécurité sociale et de 800 millions d'euros des administrations publiques locales

de plus de 5 milliards d'euros et d'une hausse importante de ses recettes, grâce au niveau de croissance inattendu en 2017. En réalité, il faut le dire, les dépenses de l'État ont fortement dérapé au cours de l'année 2017, puisque les dépenses des ministères augmentent à un niveau jamais vu depuis dix ans, avec une hausse de plus de 4 %, soit plus de 9 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. peut s'expliquer, en partie, par les nécessaires abondements de certains budgets, elle est aussi liée à un certain nombre de mesures catégorielles : je pense notamment à l'augmentation du coût des mesures « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » et du dégel du point d'indice des fonctionnaires sur les dépenses de personnel, qui représente tout de même 3 milliards d'euros en 2017. Les dépenses de personnel ont ainsi augmenté de près de 4 points l'an passé, soit plus qu'au cours des six dernières années cumulées. Avec la reprise des dépenses d'investissement, nécessaires à la croissance, cette hausse imposée des dépenses de personnel explique plus de 90 % de la hausse de 1,5 point des dépenses des administrations locales en 2017.

L'intégration, dans l'objectif maximal d'évolution des dépenses publiques, des mesures catégorielles, normes ou dépenses imposées par l'État aux collectivités territoriales est inique, L'objectif de dépense, inflation comprise, sera très difficile à tenir, et le malus qui sera alors automatiquement appliqué va, une nouvelle fois, porter atteinte aux finances des collectivités, déjà durement malmenées ces dernières années, tandis que l'application du bonus,

Comme d'autres, nous choisissons l'abstention. Surtout, comme d'autres, nous invitons le Gouvernement à prendre le taureau par les cornes et à s'attaquer vraiment à la réduction de la dépense publique pour l'exercice qui est devant nous. La parole

avec ce débat, nous allons enfin pouvoir non pas solder les comptes du quinquennat de François Hollande- ce serait trop beau et trop simple ! -, mais en tourner la page et porter une appréciation sur la première année de ce nouveau quinquennat. Que dire du dernier budget adopté par l'ancienne majorité, pour ne pas être trop cruel ? Qu'il fut, à l'image du quinquennat, une somme de contradictions,

Que nous reviendrions sous les 3 % de déficit en 2013, que nous atteindrions l'équilibre budgétaire en 2015 et que l'inversion des courbes du chômage et de la dette se produirait en 2013 ou 2014. Rien de tout cela n'est advenu, cher Claude Raynal ! C'est en

pendant que certains s'en disputaient la paternité, les uns revendiquant le fruit tardif de la politique de la majorité sortante et les autres invoquant l'enthousiasme suscité par l'élection du nouveau Président de la République, les indicateurs se sont assombris, sur fond d'une guerre commerciale qui pourrait avoir de lourdes conséquences. En même temps, le Gouvernement multipliait les annonces de dépenses nouvelles : suppression complète de la taxe d'habitation- certes, le Conseil constitutionnel y pousse, mais son financement pose question

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui du projet de loi de règlement pour l'année 2017 et de l'orientation de nos finances publiques. Cette discussion générale conjointe est particulièrement bienvenue. En effet, l'examen du passé permet d'éclairer l'avenir, même si celui-ci manque singulièrement de précision cette année, faute d'éclairages détaillés du Gouvernement sur les grandes options qu'il pourrait retenir pour le projet de loi de finances pour

La France est ainsi parvenue, pour la première fois depuis 2007, à passer sous la barre des 3 % du PIB, donc à sortir de la procédure pour déficit excessif, ouverte à son encontre au plan européen depuis 2009.

Le Gouvernement met en valeur ses efforts en matière de dépenses pour tenir compte de l'audit quelque peu alarmiste que la Cour des comptes a réalisé en juin 2017. La vérité est que la réduction de nos déficits publics s'est poursuivie de manière aussi constante qu'ininterrompue depuis 2012, année où l'on enregistrait encore un déficit de 5 % du PIB. Eh oui ! Toute la question est désormais de savoir si ce mouvement se poursuivra, et avec quelle ampleur, alors même que la conjoncture économique, quoique fragile, est aujourd'hui bien plus porteuse que celle des années passées pour améliorer la situation de nos finances publiques. Nous disposons désormais, grâce au projet de loi de règlement, d'une photographie très précise de l'exécution des comptes de l'État en 2017. Cette photographie a permis à la commission des finances d'identifier, en toute indépendance, les missions sur lesquelles une audition du ministre en exercice lui semblait la plus nécessaire, en complément des auditions qu'elle réalise tout au long de l'année. Nous avons ainsi entendu Mme Muriel Pénicaud et M. Stéphane Travert sur l'exécution de leurs crédits budgétaires. Pour éclairantes qu'elles soient, et il faut en remercier les ministres, ces auditions ont surtout permis de confirmer les constats, sans permettre d'anticiper sur les arbitrages à l'oeuvre pour les prochaines lois de finances.

qu'ils ont pu mener ces derniers mois. Je ne doute pas que le Gouvernement, particulièrement attentif à nos travaux de contrôle, en fera le meilleur usage. Le rapport compte, en effet, pas moins de 586 pages. Ce contrôle de l'exécution n'aura de sens que s'il alimente le débat et les amendements sur le projet de loi de finances, qui, rappelons-le, est l'acte juridique par lequel le Parlement consent à l'impôt et autorise la dépense publique. la photographie offerte par le projet de loi de règlement du budget de l'État n'est pas suffisante pour nourrir le débat budgétaire. Tout d'abord, elle ne saisit qu'une partie du paysage de nos finances publiques.

Il conviendrait d'élargir le champ de ce contrôle en exécution, pour le rendre plus pertinent. Ensuite, le débat sur l'exécution intervient trop tardivement, à la mi-juillet, alors même que le Gouvernement est engagé depuis longtemps dans la préparation du budget 2019. Il devrait avoir lieu au printemps, pour peser véritablement sur les choix de l'année suivante. Un effort devrait être réalisé afin de clore les comptes et de les présenter au Parlement Enfin, malgré son caractère tardif, ce débat sur l'exécution ne s'accompagne pas du dévoilement des projets et des intentions du Gouvernement, alors même que ceux-ci devraient être soumis au débat parlementaire

Dans son discours devant le Congrès, lundi dernier, le Président de la République a indiqué : « le Premier ministre présentera dans quelques semaines les nouvelles décisions permettant de tenir les engagements de baisse de nos dépenses publiques prises devant les Français. » président, il a renvoyé les décisions les plus importantes après le dépôt du projet de loi de finances, en indiquant que « d'ici à la fin de l'année, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions pour la transformation indispensable de l'action publique. Mes chers collègues, ma conviction est que, à l'heure où le Gouvernement souhaite accélérer le temps parlementaire, une plus grande transparence sur ses choix budgétaires serait profondément bienvenue.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, bien qu'il soit défini comme une étape dans la préparation du projet de loi de finances à venir, le débat d'orientation des finances publiques permet, en principe, l'examen par le Parlement des perspectives des finances publiques pour l'ensemble des administrations publiques. En théorie, il permet ainsi le suivi, année après année, des trajectoires tracées par la loi de programmation des finances publiques. En théorie également, il offre une vision complète de la contribution des administrations de sécurité sociale, qui intéresse particulièrement notre commission, aux résultats de nos comptes nationaux. Or que nous apprennent concrètement les dix lignes de bilan et la page de perspectives

de solidarité vieillesse, le FSV, s'est réduit, à 5 milliards d'euros, ce que nous savons depuis la mi-mars. L'unique page que le rapport consacre aux perspectives nous annonce, quant à elle, une refonte des exonérations ciblées, la suppression de certaines taxes à faible rendement ou encore la poursuite de la rationalisation des niches sociales, et rappelle les principaux items du plan ONDAM 2018-2022. Nous n'en saurons pas plus sur l'impact attendu de ces différentes mesures sur la trajectoire des comptes sociaux ... Pour qui s'intéresserait, par exemple, à l'évolution des dépenses d'assurance chômage- près de 40 milliards d'euros -, au résultat des hôpitaux- moins 1,5 milliard d'euros -ou encore au détail des 226 milliards d'euros de la dette sociale, la déception menace.

Quant à la supposée rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, dix lignes- dix lignes, que le Gouvernement remettra un rapport au Parlement, rapport dont le délai de remise était fixé au premier trimestre par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022. Nous resterons, là aussi, avec nos interrogations. Je rappelle que l'intégration, dans la trajectoire des administrations de sécurité sociale, les ASSO, de la révision des règles de compensation à la sécurité sociale des allégements de cotisations, qui est la traduction de ce que le Gouvernement entend par « rénovation des relations entre l'État et la sécurité sociale », avait justifié, pour notre commission, le rejet de cette trajectoire dans la loi de programmation des finances publiques. Dans le cadre du raisonnement « toutes administrations publiques », pourtant défendu par le Gouvernement, il n'a pas semblé rationnel à votre commission des affaires sociales de transférer à l'État des excédents

Je rappelle ainsi que, à la différence du budget de l'État, les régimes d'assurance sociale sont financés par des recettes affectées, ce qui répond à leur logique propre. On peut, par exemple, expliquer aux Français qu'il faut augmenter leurs cotisations de retraite, parce que le régime est en déséquilibre ; c'est d'ailleurs ce qui a été fait ces dernières années. Nos compatriotes comprendraient moins que cet effort doive être consenti au profit de la réduction du déficit du budget de l'État. C'est toute la différence, qui reste pertinente, entre un impôt et une cotisation. Or il nous apparaît que ces deux notions subissent un brouillage croissant au sein même des différents projets du Gouvernement. Pour la réforme annoncée des retraites, le slogan « un euro cotisé ouvre les mêmes droits » est une parfaite illustration de la spécificité de la notion de cotisation sociale et d'une évolution vers un schéma de financement purement contributif. le financement de l'assurance chômage s'éloigne d'un modèle assurantiel pour des raisons qui n'ont pas été explicitées au-delà de l'objectif d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Peine perdue : les Français n'auront retenu que l'augmentation de la CSG Nos compatriotes peuvent consentir à la CSG comme impôt de la sécurité sociale, en particulier comme impôt de l'assurance maladie. Il ne me semble pas que ce soit la bonne recette pour l'assurance chômage qui reste une assurance contre la perte de revenus.

cela fait beaucoup de « pognon » ! - ne donnent pas lieu à plus de détails. J'y vois, malheureusement, les effets d'un examen conjoint des différents secteurs des administrations publiques et l'illustration du besoin d'un rendez-vous parlementaire plus structuré sur le bilan et les perspectives des comptes sociaux. Je vous remercie

et ceux que nous vous proposons. Le débat budgétaire pourra d'ailleurs changer certains éléments, si vous le souhaitez. Ces plafonds sont conformes à la loi de programmation des finances publiques et à l'autorisation de transparence et d'engagement qu'a consentie le Parlement au Gouvernement. En quoi consiste un débat d'orientation des finances publiques ?

nous ne renonçons pas aux recettes des années précédentes, ni à celles qui sont en cours- c'est au ministre de l'économie et des finances qu'il revient de présenter la mesure fiscale proposée par le Président de la République. Nous renonçons aux recettes futures,

Je vous remercie

nous avons examiné dans le Grand Ouest, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, l'exécution du contrat de plan pour ce qui concerne les questions d'aménagement du territoire. Qu'observe-t-on ? Nous sommes aux deux tiers de la période contractuelle 2014-2020. Pourtant, moins d'un tiers

29 % des contrats de travail signés par des jeunes en début d'année sont des contrats d'un jour. Vous allez les faire rêver, en leur disant que l'on passe de 35 heures Un tiers des jeunes, quelle que soit la sensibilité politique de leurs parents, ont un contrat d'un jour. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans leur tête ?

mais aussi de faciliter la vie des usagers et, en même temps, d'améliorer les conditions de travail des agents. Il n'y a pas forcément d'opposition entre les conditions de travail des agents, les économies et le rôle des usagers. Vous avez présenté, monsieur le ministre, avec Mounir Mahjoubi, dix-sept premiers projets

Le scrutin est ouvert.

La séance est reprise.

vous m'ôtez les mots de la bouche. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription de la suite de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel à l'ordre du jour du lundi 16 juillet le matin, l'après-midi et, éventuellement, le soir, à la suite de la discussion générale sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ainsi que de l'examen de la proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges.

J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein d'éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion,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 Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein

en matière de gestion de l'apprentissage. C'est assez étonnant et à contre-courant de ce qu'il convient de faire. J'ajoute que l'on va confier cette gestion aux filières, en particulier aux branches.

une partie de la représentation socio-professionnelle, en particulier le patronat, refuse de signer des conventions ou laisse les conventions actuellement en vigueur, notamment les conventions de branche, arriver à leur terme sans signer de

dotée de la personnalité morale chargée notamment de répartir les financements, d'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts, de contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées, d'établir le répertoire national des certifications professionelles, d'émettre des recommandations et de mettre en oeuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage. Cette variété de missions s'explique par le fait que France compétences résultera

que cette fusion ira dans le sens d'une simplification, tel n'est pas notre avis. Cette multitude de missions confiées à France compétences montre au contraire, à nos yeux,

Mme Cathy Apourceau-Poly. La création d'un organisme national chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage En effet, alors que 97 % des organismes de formation sont à but lucratif, il est légitime que l'État veille à ce que les formations proposées ne répondent pas à la seule logique de la rentabilité et du moindre coût, au détriment de la qualité. Toutefois, plusieurs doutes persistent sur la forme que devra prendre cette instance. Premièrement, la disparition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pose la question de la participation des organisations syndicales. En effet, le rôle central que les partenaires sociaux jouent actuellement dans ces structures témoigne d'une particularité de notre modèle social

ceux des employeurs, l'État et les collectivités territoriales, il est essentiel d'assurer à cette multitude d'acteurs une place importante. C'est l'un des enjeux de cet amendement : assurer un équilibre des pouvoirs au sein de l'équipe statutaire et renforcer les pouvoirs du conseil d'administration. En effet, la nomination des personnalités qualifiées sur la seule initiative du ministère ne peut conduire qu'à donner une majorité à l'État au sein de ce conseil d'administration.

tout service public est présumé avoir un caractère administratif et confère donc un statut d'établissement public administratif à sa structure organisatrice. L'amendement n° 571 rectifié, présenté par

Il importe donc de déterminer les éléments qui seront pris en compte dans la répartition des fonds alloués aux régions : nombre d'apprentis, de CFA et de sections d'apprentissage, information sur la population. En effet, il apparaît d'ores et déjà que les fonds alloués aux régions au titre de la péréquation

Il s'agit d'éviter de donner l'avantage aux centres de formation déjà suffisamment dotés, là où la démographie est forte, et d'assurer un rééquilibrage en direction des territoires ruraux et semi-ruraux, afin d'éviter que les établissements accueillant moins d'élèves ne soient condamnés, renforçant ainsi la fracture territoriale. L'amendement

Mme Jacky Deromedi. Le projet de loi prévoit la disparition de la Commission nationale de la certification professionnelle et son remplacement par une commission de la certification professionnelle intégrée à France compétences. La disparition de la procédure indépendante et transparente de certification met en danger la crédibilité des titres enregistrés sur demande, notamment par les organismes privés d'enseignement et de formation professionnels : elle remet en cause le principe même de l'indépendance des décisions prises par la CNCP depuis 2002,

nous proposons le maintien de la CNCP, qui est responsable de l'établissement du répertoire national des certifications professionnelles, de l'inventaire et du cadre national des certifications, sans tutelle de France compétences sur ses décisions d'enregistrement ; nous souhaitons en outre la doter des moyens juridiques de son indépendance et de son fonctionnement.

La commission n'est pas non plus favorable à ce que les agents de cette agence relèvent du droit public, et considère qu'il n'est pas logique de prévoir un avis conforme du conseil d'administration sur la désignation d'une partie de ses membres.

Or la rédaction proposée fait obstacle à ce que d'autres critères soient ajoutés à ceux qui sont cités, par exemple des critères relatifs aux ressources des conseils régionaux, à l'économie régionale et à ses besoins. J'invite néanmoins Mme la ministre à nous confirmer que ces dimensions seront bien prises en compte.

auteurs de cet amendement plaident pour le maintien de la Commission nationale de la certification professionnelle. Toutefois, l'alinéa qu'ils proposent de supprimer se borne à mentionner que France compétences est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. La suppression de cet alinéa ne satisferait pas l'objectif des auteurs de cet amendement et créerait un vide juridique s'agissant de la gouvernance de France compétences. À moins qu'il ne soit retiré, la commission émet donc un avis défavorable sur cet le projet de loi prévoit que les agents de France compétences seront régis pas les dispositions du code du travail, y compris en ce qui concerne les relations collectives de travail. Des accords collectifs pourront donc être conclus sans qu'il soit nécessaire de le préciser explicitement dans la loi.

de la qualité des actions de formation, nous mettons pour la première fois en place une certification obligatoire de tous les organismes de formation en France qui travaillent sur fonds mutualisés

la régulation, la qualité, l'offre, la prévisibilité et le pilotage des formations. Il n'y a pas une seule compétence régionale qui irait à cette instance,

M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à corriger une formulation inadéquate : le fonds pour le financement des centres de formation des apprentis n'est pas à proprement parler un mécanisme de péréquation territoriale ; il s'agit d'un montant dont l'usage est librement déterminé par les régions. Quel

Depuis 2015, ils ont la possibilité d'accéder au service public régional de la formation professionnelle. Ce dispositif est très utile, car il permet, notamment, d'apporter une solution aux expatriés qui envisagent une réinsertion professionnelle en France, mais qui n'ont pas la possibilité de bénéficier de formations dans leur pays de résidence. Chaque année, entre soixante et quatre-vingts personnes bénéficient de ce dispositif, dont les modalités ont été précisées par une convention conclue en mars 2015 entre le ministère des affaires étrangères, le ministère du travail, Pôle emploi et l'Association des régions de France. En vertu de cette convention, les postes consulaires assurent le premier accueil des candidats et transmettent les demandes de formation à Pôle emploi. Ce dernier organisme offre des prestations d'orientation, d'organisation du parcours de formation et de suivi personnalisé. Quant aux régions, elles sont chargées du financement des actions de formation et de l'hébergement, ainsi que du bilan et de l'évaluation du parcours de formation. Afin de parachever l'intégration des Français établis hors de France dans le droit commun de la formation professionnelle, nous proposons de confier à France compétences la mission de suivre l'application de la convention du 18 mars 2015. L'évaluation de la qualité des prestations offertes à nos concitoyens résidant à l'étranger permettra notamment à France compétences de formuler, en tant que de besoin, des recommandations en vue d'améliorer le dispositif prévu à l'article L. 6121-2 du code du travail.

Il prévoit en outre que l'État, les régions et les partenaires sociaux pourront lui en confier d'autres. Afin de ne pas allonger inutilement la loi et de laisser au conseil d'administration et au directeur général une certaine marge d'appréciation dans la gouvernance de l'agence,

de handicap et de leurs besoins importants en matière de formation professionnelle, il apparaît nécessaire d'ajouter une mission à l'établissement public France compétences que crée l'article 16 de ce projet de loi. L'ajout de cette mission doit permettre le renforcement de l'accès à la formation professionnelle et à l'apprentissage des travailleurs en situation de handicap. Par ailleurs, France compétences doit également être en mesure d'établir des recommandations sur l'accès des travailleurs handicapés à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, de manière à s'assurer que cette mission est pleinement incluse dans les missions de l'établissement public et qu'elle constitue ainsi un sujet de préoccupation réelle.

? Je ne suis pas certain qu'une telle disposition ait réellement une portée normative. En effet, qu'est-ce qui définit un travail d'observation validé scientifiquement ? Interprété strictement, cette disposition contraindrait de manière excessive les recommandations que France compétences sera en mesure de formuler. On peut même se demander si, dans certains domaines des politiques publiques, une démarche scientifique est réellement possible. Des constats et des recommandations peuvent être valides sans que les travaux qui y mènent soient nécessairement qualifiés de scientifiques. Je pense notamment aux travaux de contrôle que nous produisons dans cette institution. La commission demande donc le retrait

de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Les dispositions du projet de loi prévoient la communication à France compétences de certaines données, notamment par la Caisse des dépôts et par les et par les opérateurs de compétences. Il ne me semble donc pas utile de préciser que France compétences a le droit de traiter ces données transmises dans un cadre officiel.

et par le titre XIII de la Constitution. Si ces collectivités en font la demande, un partenariat pourrait être noué entre les instances en charge de la formation professionnelle au sein de ces collectivités et le nouvel organisme France compétences. Ce partenariat permettrait d'assurer le développement de la formation professionnelle sur ces territoires, mais aussi l'articulation des politiques menées en matière de formation professionnelle par la France et les différentes collectivités d'outre-mer. Quel

mais ne saurait constituer une mission en tant que telle. Au demeurant, la rédaction de cet amendement ne précise ni le contenu ni l'objet de ces conventions. En outre, conformément à la position que j'ai exprimée sur d'autres amendements, la commission n'est pas favorable à ce que la liste des missions de France compétences soit davantage élargie,

France compétences doit être un lieu de gouvernance quadripartite associant l'État, les régions et les partenaires sociaux. Il n'est pas souhaitable de faire entrer au sein de son conseil d'administration toute une série d'autres acteurs. Si l'on adoptait l'ensemble des propositions formulées par les uns et les autres, le conseil d'administration de France compétences comprendrait, outre l'État, les régions, les organisations syndicales et les organisations patronales, des représentants des départements, des communes, du secteur de l'inclusion, des organismes consulaires, des établissements certificateurs et des associations représentant les personnes handicapées, les personnes précaires et les demandeurs d'emploi. Je vous laisse imaginer à quoi il ressemblerait Cette énumération donne une idée de la taille qu'aurait alors le conseil d'administration et l'on comprend à quel point cette agence serait ingouvernable, devenant rapidement inutile. De plus, si l'État, les régions et les partenaires sociaux sont parties prenantes de l'ensemble des missions confiées à France compétences, les acteurs visés à ces amendements

chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation puissent participer à la désignation des cinq personnalités qualifiées qui siégeront au sein

classent les offres pour le conseil en évolution professionnelle avant que France compétences ne choisisse l'opérateur. Le cahier des charges sera bien établi de façon quadripartite- État,

Plusieurs dispositions du texte prévoient déjà des obligations de transmission à France compétences. En outre, le décret d'application dont le présent amendement vise à préciser le contenu doit fixer les conditions d'application de la section relative à France compétences

Sa répartition et ses bénéficiaires sont-ils appelés à être modifiés ? La commission a adopté un judicieux amendement qui tend à exclure les établissements d'enseignement supérieur à but lucratif de la liste des potentiels bénéficiaires. En revanche, la question de la répartition de ces fonds suivant les niveaux de formation reste posée. Aujourd'hui, cette répartition est obligatoirement de 65 % pour la catégorie A et de 35 % pour la catégorie B. Est-il envisagé une nouvelle répartition ?

Cette décision n'est pas neutre pour les lycées professionnels privés sous contrat avec l'État qui participent au service public de l'éducation par leur association avec l'État. Pour autant, ces établissements n'ont pas les mêmes ressources que les lycées professionnels publics. Il serait donc souhaitable que, durant nos débats, vous nous indiquiez vos intentions sur les possibilités d'une modulation du coût des contrats en fonction des ressources publiques permettant de préserver ces établissements, très présents sur certains territoires et dans diverses activités.

Dans sa rédaction initiale, le Gouvernement prévoyait la fusion de la taxe d'apprentissage et des contributions au financement de la formation professionnelle, ainsi que la création d'une contribution unique au financement de la formation professionnelle et de l'alternance, collectée par les organismes de sécurité sociale- le réseau des URSSAF notamment -et affectée à France compétences chargée de la répartir. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, les députés de la majorité sont revenus sur cette rédaction, de telle sorte que les changements concernent uniquement la collecte des contributions réalisée par les URSSAF et l'affectation de leur produit à un organisme unique. Le financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage est un sujet crucial pour l'avenir de notre pays, notamment face à la transition numérique. Les besoins de formation vont être croissants et, pour y répondre, nous devons augmenter les ressources de la formation. En tant que parlementaires, nous ne pouvons débattre d'une réforme du système de financement de la formation

les taux actuels s'agissant de la taxe d'apprentissage comme des contributions des entreprises au développement de la formation professionnelle. Il ne me semble donc pas justifié d'affirmer que la contribution financière des entreprises serait réduite.

par l'URSSAF aux opérateurs de compétences qui financent directement les contrats en alternance, sans transiter par France compétences, qui n'a pas de valeur ajoutée en la matière. Les opérateurs de compétences sont soumis à des délais de règlements de trente jours maximum à compter de la réception des justificatifs de réalisation, le non-respect de ces délais étant considéré comme une défaillance pouvant entrainer la nomination d'un administrateur provisoire de l'opérateur. Ainsi, l'étape France compétences emporte un risque de tension de trésorerie et, en conséquence, d'allongement du délai de paiement, ce qui serait préjudiciable aux organismes de formation et aux CFA.

collectés par les URSSAF pour le financement de la formation professionnelle et de l'alternance. Prévoir que les URSSAF opèrent une première répartition de ces fonds entre France compétences et les opérateurs de compétence, alors même que France compétences versera par ailleurs aux OPCO les sommes destinées au financement du développement des compétences, complexifie inutilement le circuit

Mme Jacky Deromedi. Le projet de loi oblige les entreprises à affecter directement une partie de leur taxe d'apprentissage à des établissements et organismes dûment habilités, mais ne prévoit rien en cas de non-affectation. Dans ce cas, le risque est double : d'une part, que le comptable de l'entreprise verse sa taxe au Trésor public que, faute de contrôle, il ne verse rien. Dans les deux cas, cette part de fonds non affectés, dite « fonds libres », échappe aux établissements dûment habilités. Afin d'éviter ce risque d'évaporation, cet amendement tend à sanctuariser ces fonds libres par un versement des fonds non affectés aux URSSAF, qui en confient la gestion

de la commission ? Les dépenses prévues au titre du solde de la taxe d'apprentissage n'auront pas à être affectées par les entreprises comme c'est le cas actuellement pour le « hors quota

générale des finances publiques, dans la période transitoire. Toutefois, nous souhaitons privilégier cette relation directe entre l'entreprise et l'établissement bénéficiaire, car nous savons par expérience que c'est le gage d'une meilleure relation entre entreprises et établissements d'enseignement pour la partie «

dispositions de cet amendement résultent d'un malentendu fortement lié à l'improvisation qui semble entourer la réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par l'article 17. En effet, cet article a été intégralement réécrit par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement. Cette réécriture en cours d'examen n'a pas permis qu'une étude d'impact sérieuse soit réalisée, ni que la rédaction proposée soit soumise pour avis au Conseil d'État. C'est regrettable, compte tenu des sommes en jeu. Par ailleurs, les explications fournies dans le rapport de nos collègues de l'Assemblée nationale sont relativement laconiques, et celles que le Gouvernement a apportées à nos collègues dépités en séance publique n'ont guère permis de mieux comprendre l'opération. Aujourd'hui, la fraction de la taxe d'apprentissage destinée au « hors quota » représente 23 % du produit de cette taxe. Toutefois, une partie substantielle de ce « hors quota » est affecté à des CFA en complément des sommes versées au titre du quota. Dans les faits, en 2016, les établissements éligibles au « hors quota » ont reçu 14,2 % du produit de la taxe d'apprentissage. Or, avec la réforme proposée, l'intégralité du solde de la taxe d'apprentissage sera attribuée à ces établissements, sans possibilité de reversement aux CFA. Compte tenu des prévisions d'évolution de la masse salariale, à horizon de 2020, lorsque la réforme prévue par l'article 17 sera effective, quelque 13 % du produit de la taxe d'apprentissage permettraient aux établissements concernés de recevoir une masse financière équivalente, voire supérieure en valeur, à celle qu'ils reçoivent aujourd'hui. Il y a donc une légère baisse en volume, mais sans que celle-ci atteigne l'ampleur que craignent les auteurs de l'amendement. Fixer le solde de la taxe d'apprentissage à 23 % constituerait donc une augmentation considérable des sommes affectées aux établissements éligibles, au détriment des CFA.

Merci